L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires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

La distinction entre la détention légitime et l'obtention licite du secret est conservée, alors que le texte initial confondait les deux notions, du fait d'une certaine méconnaissance de la directive transposer. La clarification de la rédaction des cas d'obtention illicite est maintenue, en conformité avec la directive. Le caractère « non opposable » du secret des affaires- plutôt que « non protégé

Sur ce point, le juge devra tenir compte des travaux préparatoires dans son office d'interprétation de la loi. L'amende civile en cas de procédure abusive, introduite par l'Assemblée nationale,

en matière constitutionnelle : nous avions introduit un élément matériel précis, à savoir le contournement délibéré des mesures de protection destinées à conserver le caractère secret de l'information.

été quintuplée pour une personne morale, par application des règles de droit commun : ce serait plus efficace, compte tenu des personnes visées. D'autre part, on pourrait prévoir sans trop de difficulté

a pour objet de clarifier les différentes étapes de la procédure par laquelle un juge peut être amené à décider de mesures particulières de protection du secret des affaires concernant une pièce discutée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans un premier temps, le juge examine seul la pièce pour décider si la demande de protection au titre du secret des affaires est justifiée. Éventuellement, avant de rendre sa décision, il peut demander une expertise et solliciter l'avis des seuls avocats des parties, ceux-ci étant tenus dans ce cas à une obligation de confidentialité vis-à-vis de leurs clients. Dans un second temps, le juge décide s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection.

Je tiens à mon tour à saluer la manière dont, sur un sujet difficile et complexe, vous avez su trouver des voies de passage et inventer des équilibres subtils dans un cadre européen très contraint. Vous avez aussi su répondre aux interrogations, nombreuses, qui se sont fait jour dans les médias et l'opinion sur ce texte. Ces questions étaient légitimes

La rédaction adoptée par la commission mixte paritaire garantit ce respect. Les termes employés, qui sont ceux de la directive, ne donneront pas lieu à d'inutiles polémiques sur le champ de la protection accordée au secret des affaires. Il est bien clair, désormais, que toutes les données de nature économique détenues par une entreprise ne peuvent être qualifiées de « secret des affaires ». Seules le seront celles qui font l'objet de mesures raisonnables de protection et qui revêtent une valeur commerciale, effective ou potentielle, pour leur détenteur. Ce dernier devra en rapporter la preuve. Un second point était en discussion : l'introduction d'une nouvelle sanction pénale pour « détournement d'une information économique protégée Le Gouvernement n'y était pas favorable. J'avais eu l'occasion de l'indiquer ici même et nous en avions débattu. La transposition de la directive ne l'imposait pas, le législateur européen ayant fait le choix, clairement assumé, d'un dispositif uniquement civil. Nous avions également une divergence d'appréciation sur la définition de ce délit et sa précision. Pour autant, les préoccupations exprimées étaient justes : nos entreprises doivent disposer des moyens de se défendre contre l'espionnage industriel, dans un contexte de mondialisation et de concurrence exacerbée, qualifiée de « guerre économique » par votre rapporteur.

et Gauvain une mission afin que soient analysées les mesures juridiques de protection des entreprises françaises confrontées à des procédures judiciaires ou administratives de portée extraterritoriale. Dans ce cadre, on pourra notamment évaluer l'intérêt d'une réforme de la loi du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage », relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. Enfin- dernier sujet d'importance -, il était selon moi particulièrement opportun que la commission mixte paritaire maintienne la disposition sur l'amende civile introduite par le député Raphaël Gauvain, afin de répondre aux vives préoccupations exprimées quant au risque de « procédures bâillons ». J'avais bien entendu les interrogations de votre rapporteur sur la pertinence et même la constitutionnalité de ce dispositif. Nous en avions débattu de ce dispositif. Nous en avions débattu dans cet hémicycle. Mais rappelons simplement que cette mesure a pour objet de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner des procédures abusives qui, en la matière, peuvent porter une atteinte particulièrement forte à l'exercice du droit fondamental à la liberté d'expression. Je suis convaincue que cette disposition constituera un outil efficace et équilibré de préservation et de protection des droits fondamentaux, à l'occasion des actions conduites aux fins de prévention, de cessation ou de réparation d'une atteinte à un secret des affaires. Les journalistes et lanceurs d'alerte ne peuvent pas et ne doivent pas faire l'objet de poursuites judiciaires exclusivement fondées sur une volonté d'intimidation. L'objectif poursuivi au travers de cette proposition de loi n'est certainement pas, comme j'ai pu l'entendre et le lire, de restreindre la protection juridique accordée aux lanceurs d'alerte ou de porter atteinte à la liberté de la presse. Ce texte n'a nullement pour objet de rendre impossible le journalisme d'investigation, ni pour effet d'empêcher la révélation au grand public de faits légalement ou moralement condamnables. Je l'ai déjà dit, et je le redis ici avec la même force et la même conviction : le texte qui vous est présenté ne constitue en aucune manière un recul pour les libertés publiques. L'enjeu est bien de protéger les entreprises contre le pillage de leurs innovations. Il est aussi de lutter contre la concurrence déloyale. Il consiste encore à encourager la recherche et le développement, sources de nombreux emplois. Pour cela, les acteurs économiques ont à l'évidence besoin de sécurité juridique. C'est le seul objectif de cette proposition de loi : définir les informations qui relèvent du secret des affaires et encadrer les demandes formées devant le juge pour la protection de ce secret.

Les juridictions y veilleront. Ainsi, une entreprise ne pourra pas se prévaloir d'un secret des affaires pour s'opposer aux enquêtes judiciaires ou administratives dont elle ferait l'objet. Elle ne pourra pas davantage s'opposer à la révélation d'un secret des affaires lorsque cette révélation est nécessaire pour l'exercice d'un droit syndical. Elle ne pourra pas non plus obtenir du juge qu'il empêche la diffusion au grand public d'une information d'intérêt général au motif que cette information constituerait un secret des affaires. Elle ne pourra pas, enfin, obtenir des dommages et intérêts d'un salarié qui, de bonne foi et dans un but d'intérêt général, a porté à la connaissance d'un journaliste une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. En cas de révélation d'un secret des affaires, journalistes et lanceurs d'alerte pourront toujours se prévaloir d'avoir agi dans le dans le cadre de l'exercice légitime de leur liberté d'expression et d'information. Ces principes sont très clairement et très heureusement énoncés dans la présente proposition de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est aujourd'hui soumis, fruit de réflexions approfondies menées depuis plusieurs années, constitue selon moi une réelle avancée de notre système juridique. Cette amélioration a été construite sans que soit portée pour autant une atteinte injustifiée aux droits fondamentaux et au cadre juridique protecteur des lanceurs d'alerte. Protéger le secret des affaires est devenu une nécessité.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous allons adopter est une réponse juridique à la nécessité de protéger l'intelligence économique européenne.

des comportements internationaux, en particulier outre-Atlantique, évolution qui nous pose des problèmes particuliers. À mon sens,

Pour tout vous dire, madame la ministre, ce sujet n'est pas inconnu de cette maison : la commission des affaires européennes avait fait le choix, il y a quelques mois, de travailler sur cette question, et nous présenterons dans quelques jours nos propositions. Je ne vous cacherai le sujet est complexe ; plus exactement, le caractère opérationnel des mesures que nous pourrions proposer n'est pas aisé

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quand les visiteurs du Palais du Luxembourg passent dans la salle du Livre d'or, ils y apprennent que les fenêtres, d'époque, doivent beaucoup à un espionnage industriel mené aux dépens des cités-États italiennes, qui maîtrisaient le secret de la fabrication du verre ... Oui, l'espionnage industriel a toujours existé, il a toujours été combattu, et le groupe socialiste et républicain est évidemment attaché à défendre les savoir-faire de nos entreprises dans la compétition acharnée qui se joue à l'échelle mondiale.

Y avait-il une telle urgence à transposer la directive européenne, alors que seul le Danemark l'a fait à ce jour ? Fallait-il user d'une procédure accélérée ?

alors même que s'annonce une proposition de résolution européenne sur les lanceurs d'alerte, qui pose dans des termes différents nombre des questions que nous avons dû traiter sur le secret des affaires Notre collègue François Pillet nous indiquait d'ailleurs hier que « la proposition de directive ne prévoit aucune articulation particulière avec l'exception à la protection du secret des affaires prévue au bénéfice des lanceurs d'alerte par la directive » » et que « l'existence dans le droit européen de deux régimes distincts serait une source de complexité et de confusion. » Vous l'avez constaté comme moi, sur ce texte, la précipitation a été mauvaise conseillère. Notre seconde réserve tient évidemment au fond. Plusieurs inquiétudes de nature différente ont été exprimées au sujet de cette proposition de loi. Des doutes subsistent encore aujourd'hui sur ses conséquences juridiques, malgré les évolutions issues des travaux de la commission mixte paritaire. une certaine imprécision s'agissant de la définition du champ exact des informations protégées, des atteintes possibles à la liberté d'expression ou,, de possibles oppositions entre le droit de la presse et le droit commercial, ainsi que des restrictions au droit de participation des travailleurs. Je devine que ces arguments n'ont pas porté de la même manière selon nos positions dans cet hémicycle ! S'ils ne pèsent pas suffisamment aujourd'hui, ils trouveront peut-être plus d'écho dans d'autres lieux de délibération de la République, car les sénateurs socialistes ont choisi de déposer, si ce texte est voté, un recours devant le Conseil constitutionnel. Cette décision n'allait pas de soi et n'est pas automatique : vous connaissez la sagesse des sénateurs, fussent-ils socialistes, et leur habituelle tempérance. Toutefois, face à l'absence de consensus sur ce texte, encore dénoncé par une alliance d'associations, de syndicats, de journalistes et de lanceurs d'alerte qui a atteint une taille critique, face aux craintes encore ressenties aujourd'hui par les centaines de milliers de citoyens qui ont exprimé leur opposition, le groupe socialiste et républicain a jugé qu'il était pertinent de solliciter une nouvelle expertise. Si la délibération parlementaire touche bientôt à sa fin, les travaux du Conseil constitutionnel éclaireront peut-être notre réflexion commune. Il y a plusieurs manières d'aborder ce débat. ce débat. Comme le rapporteur à l'Assemblée nationale, qui était avocat d'affaires jusqu'à son élection aux dernières législatives, ou nombre de partisans de ce texte dans cet hémicycle, on peut se féliciter que les entreprises obtiennent les moyens de se protéger. plusieurs représentants de syndicats ou d'associations que nous avons rencontrés ne s'en privent pas. Ils doutent notamment que ce texte serve effectivement à des PME dans le futur craindre, surtout, qu'il ne soit détourné de son objectif et ne serve à tenter de museler des lanceurs d'alerte ou des journalistes. Secret des affaires contre liberté d'informer, ce débat n'est pas secondaire Certains m'objecteront que des dispositions ont été introduites dans le texte pour éviter toute dérive, notamment des sanctions contre les « procédures bâillons ». Elles ne suffisent cependant pas à rétablir l'équilibre entre secret des affaires et liberté d'informer. Ceux qui ne sont pas Ceux qui ne sont pas convaincus par ce texte- je ne parle pas ici des parlementaires -connaissent les enjeux que nous évoquons aujourd'hui. Ils ne sont ni stupides, ni bornés, ni mal intentionnés. Ce sont bien souvent des militants qui ont démontré leur utilité pour la société en rendant publics des scandales au profit de l'intérêt général. leur parole et leur légitimité sont remises en question. Une pétition a atteint plusieurs centaines de milliers de signatures ; les vidéos qui touchent au secret des affaires font des millions de vues ; des journalistes tentent de produire des récapitulatifs pour informer le grand public en toute objectivité. Pourtant, on remet toujours en question leurs conclusions Une partie du site internet du est consacrée au décryptage de l'actualité. Il est présenté comme suit : « Les décodeurs du vérifient déclarations, assertions et rumeurs en tous genres ; ils mettent l'information en forme et la remettent dans son contexte ; ils répondent à vos questions. » Savez-vous comment le rapporteur de l'Assemblée nationale a qualifié le travail réalisé par ce site

a, certes, été amélioré- n'en déplaise à notre respectable rapporteur Christophe-André Frassa -, mais il ne parvient toujours pas à rassurer, notamment en raison d'une définition trop large des informations à protéger.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le constat est clair : dans un contexte de compétition économique internationale toujours accrue, il manque à la législation française un dispositif général et transversal de protection du secret des affaires, afin de garantir une véritable protection des informations confidentielles détenues par nos entreprises. En effet, si, pour assurer la garantie des brevets, marques et autres dessins et modèles, le droit de la propriété industrielle est efficace, il ne suffit pas à assurer la protection des nombreuses informations économiques et techniques confidentielles des entreprises. Le diagnostic Le diagnostic de la carence du droit français en matière de protection du secret des affaires est établi depuis longtemps, de sorte que les initiatives législatives pour mieux armer nos entreprises françaises exposées à la concurrence internationale n'ont pas manqué depuis 2010. Elles ont malheureusement toutes échoué à mettre en place un dispositif civil ou pénal de protection. La proposition de loi relative à la protection du secret des affaires vise à transposer en droit français la directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, dont l'objectif est d'établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d'appropriation illicite. On peut légitimement déplorer les conditions de présentation et d'examen de ce texte

la transposition de cette directive permettra à la France de se doter d'un régime de protection du patrimoine économique, technologique et informationnel de ses entreprises. Aussi, notre groupe se réjouit, d'une part, que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion soit parvenue à un accord, et, d'autre part, que le texte adopté reprenne, pour une grande part, la rédaction retenue par le Sénat. Néanmoins, nous souhaitons modérer notre position sur deux points. En premier lieu, la commission mixte paritaire a rétabli l'amende civile spécifique que nos collègues députés avaient prévue pour sanctionner les personnes qui engageraient abusivement une action relative à une atteinte au secret des affaires.

Le Sénat avait supprimé cette disposition pour deux raisons. Premièrement, l'amende civile peut être jugée contraire aux principes constitutionnels d'égalité et de légalité des délits des délits et des peines ; deuxièmement, il apparaît probable que les juges ne l'appliquent pas, au vu de leur pratique actuelle en matière d'amendes civiles pour procédure abusive. En second lieu, la commission mixte paritaire a procédé à une autre suppression, celle du délit d'espionnage économique. Cette notion avait été introduite par la commission des lois du Sénat, afin de sanctionner le détournement d'une information protégée au titre du secret des affaires à des fins exclusivement économiques, excluant de son champ les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés. Pour le Sénat, le message devait être clair : les entreprises françaises sont soumises à une véritable guerre économique, qui ne cesse de s'amplifier. Un volet pénal avait donc toute sa pertinence, avec une amende de 375 000 euros, largement supérieure à celle qui est prévue pour sanctionner le vol. Notre groupe regrette que cette notion ait été écartée et encourage vivement les deux rapporteurs du texte à tenir leur engagement de poursuivre l'étude de cette question dans le cadre d'une mission plus large, visant à mieux armer encore nos entreprises dans cette guerre. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le président de la commission des lois, Philippe Bas, l'a souligné : « un réarmement juridique de la France s'impose contre le pillage des données ! » Nous ne pouvons que souscrire à ce point de vue. Au cours des dernières années, quelque 20 % des entreprises indiquent avoir subi au moins une tentative d'appropriation illicite de leurs secrets d'affaires, et 25 % d'entre elles ont signalé un vol d'informations confidentielles.

l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi transposant la directive sur la protection du secret des affaires intervient alors que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre les États-Unis, le Canada et l'Europe, paraît s'intensifier. Les pratiques d'espionnage économique visant les entreprises françaises et européennes, qui s'ajoutent aux vulnérabilités nouvelles liées aux cyberattaques, sont plus que jamais une réalité. Pendant longtemps, les pays européens ont manqué d'un cadre juridique réellement protecteur pour leurs entreprises. Alors que les États-Unis disposent depuis la fin des années 1990 d'un puissant arsenal de lutte contre les atteintes au secret des affaires, avec en particulier la loi Clinger-Cohen de 1996, ce n'est qu'en 2016 que les dirigeants européens ont adopté la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées- soit le secret des affaires -, qui enjoint, pour la première fois, l'ensemble des États membres à instaurer un régime général de protection des secrets d'affaires et qui rend ceux-ci opposables lors de procédures contentieuses. contentieuses. Jusqu'alors, toutes les tentatives d'instaurer un tel régime général en France avaient échoué. D'après la définition générale, un secret d'affaires est une information ayant une valeur marchande, considérée comme confidentielle par l'entreprise et qui lui donne un avantage compétitif dans son secteur. La numérisation de l'économie rend la protection des secrets d'affaires encore plus cruciale. D'après une étude publiée l'an dernier dans la revue , la France est le neuvième pays au monde le plus attaqué par les cybercriminels. Toutefois, la culture de sécurité informatique y reste étonnamment peu développée. Tout se passe comme si les usagers s'en remettaient à la solidité supposée du « système » sans imaginer que leurs outils informatiques puissent faire l'objet de piratage et que leurs données personnelles ou des informations confidentielles de leur entreprise puissent être divulguées à leur insu. Néanmoins, la révélation, ces dernières années, de plusieurs scandales, comme celui du Mediator, ou des affaires LuxLeaks et « Panama Papers a sensibilisé le public à ce sujet et a engendré une grande défiance à l'égard des acteurs économiques et de la mondialisation. La mobilisation impressionnante des organisations non gouvernementales, des organes de presse ou des lanceurs d'alerte lors de l'examen de ce texte en témoigne. Malgré les délais d'examen très courts et les marges de manoeuvre limitées du législateur, la directive sur le secret des affaires continue de susciter des craintes et des oppositions, parfois excessives. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire apparaît plutôt équilibré, dans la mesure où il effectue une transposition assez stricte du contenu de la directive, en particulier en ce qui concerne la définition du concept même de secret des affaires. Du point de vue du Sénat, même plus équilibré qu'en première lecture, puisqu'il rétablit, notamment, l'amende civile en cas de procédure dilatoire ou abusive. Par ailleurs, la pénalisation de l'espionnage économique, qui a suscité de vifs débats en première lecture et dont mon groupe avait demandé la suppression, n'a pas été retenue dans la version finale, finale, car ce type d'infraction est déjà couvert par la législation sur le vol et l'abus de confiance. Enfin, la notion de valeur commerciale effective ou potentielle de l'information protégée a été préférée à celle de valeur économique, dont l'acception paraissait trop On peut encore s'interroger sur la longueur du délai de prescription- cinq ans -en matière de violation du secret des affaires, mais, globalement, ce texte offre un cadre raisonnable et conforme à nos responsabilités de législateur, dans la mesure où il s'agit, je le rappelle, d'un texte de transposition. Comme l'avait souligné notre collègue Jean-Marc Gabouty lors de la première lecture, cette transposition constitue bien une nouveauté juridique, puisque le droit français ne définissait pas jusqu'à présent le secret des affaires, même s'il y faisait souvent référence. La protection du secret des affaires est en revanche un principe inscrit depuis longtemps dans le droit anglo-saxon, aux côtés de la législation sur les marques et les brevets. Aux États-Unis,

Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mieux protéger les entreprises européennes et françaises face à des pratiques déloyales, comme on en a connu par le passé, par exemple la conception du Tupolev soviétique, tellement copié sur le Concorde qu'on le surnommait « Concordski », l'espionnage des Américains et des Chinois dans le secteur automobile, avec en particulier une offensive menée par General Motors sur Volkswagen. L'information protégée au titre du secret des affaires répondra donc aux trois critères énoncés à l'article premier : son caractère non accessible en raison de sa nature ou de sa conception, sa valeur commerciale effective ou potentielle et, enfin, le fait de faire l'objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Le texte précise également les éléments d'appréciation que le juge devra prendre en compte, notamment la nécessité éventuelle de limiter la communication de certaines informations, la formation de jugement et les modalités de publication de la décision. La liberté d'expression et de communication reste totalement protégée par la Convention européenne des droits de l'homme comme par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Les lanceurs d'alerte, quant à eux, bénéficient d'un statut à part entière depuis la loi Sapin II de 2016. Par ailleurs, la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises a été abordée dans la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et devrait de nouveau être abordée dans le projet de loi PACTE, que nous examinerons cet automne. En résumé, ce texte doit assurer un bon équilibre entre la liberté d'information au service de l'intérêt général et la protection des connaissances à objet commercial, dans un monde économique où la naïveté n'est pas permise. D'une part, les exceptions à la protection du secret des affaires offrent des garanties aux journalistes, aux syndicats ou encore aux associations citoyennes. D'autre part,

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui, au retour d'une commission mixte paritaire conclusive, vise à assurer un niveau de protection commun du secret des affaires au sein de l'Union européenne, au profit de nos entreprises, de leur savoir-faire, de leurs innovations, contre le pillage industriel, la concurrence déloyale et ce que l'on appelle, par un euphémisme douteux, « l'intelligence économique parler franc, signifie ni plus ni moins l'espionnage économique. L'actualité récente est là pour nous rappeler de manière récurrente que ces pratiques déloyales ne cessent de se développer entre entreprises, parfois avec l'appui de services de renseignement de pays supposément alliés,

la rapporteur au Parlement européen et nous avions mis en lumière, bien avant que cela fasse polémique, le droit des journalistes et des lanceurs d'alerte, ce qui avait permis, déjà, de corriger le texte. proposition de loi n'a pas manqué d'animer les débats au sein du Parlement, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, car elle renvoie à une valeur fondamentale de nos démocraties : la liberté d'expression, pilier de nos institutions et principe fondamental de l'État de droit.

On peut, à ce titre, citer la création d'une amende civile destinée à lutter contre les « procédures bâillons » exercées à l'encontre d'un individu, d'une association ou d'une organisation et qui visent à intimider et à dissuader ceux-ci de dévoiler publiquement des informations en leur possession. Le passage au Sénat a permis d'enrichir certains aspects du texte, notamment en précisant la définition du détenteur légitime du secret et la caractérisation de l'obtention illicite du secret des affaires. Les procédures judiciaires mises en place pour garantir une protection efficace du secret des affaires ont également été clarifiées. Au fil de la discussion, le texte a toutefois été durci sur certains points, s'éloignant de l'ambition initiale de la proposition de loi et et du droit européen, avec notamment la suppression de l'amende civile pour lutter contre les « procédures bâillons » et l'insertion d'un volet pénal. L'accord trouvé en commission mixte paritaire a heureusement permis de corriger ces évolutions.

rédaction de l'article 1, qui caractérise la nature de l'information protégée par le secret des affaires, est parfaitement alignée avec la définition suggérée par la directive européenne. L'information protégée doit ainsi revêtir,

des journalistes, des lanceurs d'alerte ou des représentants des salariés s'exposeront à une amende pouvant aller jusqu'à 60 000 euros ou 20 % du montant des dommages et intérêts demandés. Enfin, l'infraction pénale insérée lors de l'examen du texte au Sénat, qui permettait de sanctionner le détournement d'une information économique protégée, a été retirée. Cette disposition n'apparaissait pas nécessaire pour répondre à l'objectif de la proposition de loi. Les travaux effectués par les rapporteurs de nos deux assemblées ont donc ont donc été utiles et méritent d'être salués, car l'accord trouvé vise bien l'objectif commun de protection des entreprises françaises contre le pillage industriel,

Cette proposition de loi a pour seul objectif de protéger, même contre l'intérêt général, toute information revêtant une valeur commerciale du fait de son caractère secret.

plus d'un demi-million de citoyens se sont mobilisés, car ce que vous proposez en guise de liberté d'informer, c'est la mise en place d'une forme de censure.

Toutes ces personnes seraient-elles à ce point dans l'erreur ? Cinquante-deux organisations feraient-elles fausse route ? Sommes-nous si nombreux à ne pas avoir compris ce texte et à surestimer les dangers qu'il comporte ? Pourtant, ainsi que nous en avons fait la démonstration lors des débats,

Vous nous répétez à l'envi que ce texte, bien entendu, ne sert qu'à protéger nos entreprises d'une concurrence féroce- et réelle -, mais vous avez refusé nos nombreux amendements qui visaient, justement, à réduire le champ d'application du secret des affaires à l'entreprise et à protéger les PME et les sous-traitants de ce secret si largement défini. Ce qui est mis en cause aujourd'hui, comme le rappelle un éminent journaliste, c'est « cette vérité qui procède de la raison par la déduction, le recoupement, la recherche, la vérification, la précision. cette vérité qui suppose l'enquête. Derrière ce mot apparemment simple, il y a un travail patient, minutieux et complexe, essentiellement collectif, où la vérité est produite, trouvée, dénichée, accouchée, débusquée ... » Cette vérité que révèlent, dans un souci de protection de l'intérêt général, en faisant fi de leur propre situation et des conséquences parfois lourdes sur leur vie personnelle et professionnelle, des chercheurs, des journalistes, des salariés, des représentants du personnel- la liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, ce que vous faites avancer, c'est la protection de l'optimisation fiscale, le chantage au fournisseur, la sous-traitance en cascade, les techniques de management douteuses, les pratiques à la limite de la légalité, mais aussi de possibles de possibles risques sanitaires et environnementaux majeurs présents et à venir : rôles des perturbateurs endocriniens, impact des pesticides sur la santé ou l'environnement, ou toute information que l'entreprise qualifiera de secrète. ne s'agit pas d'une vue de l'esprit de quelques activistes extrêmes. Aujourd'hui, de nombreux juristes dénoncent également ce texte. Deux avocats spécialisés le font en ces termes : « Imaginez que quelqu'un, au sein d'une entreprise pharmaceutique, estime qu'un produit dangereux, néfaste pour la santé ou l'environnement, a été mis sur le marché. Eh bien, la dérogation à la protection du secret des affaires serait alors probablement suspendue à l'issue d'investigations et de procédures pouvant durer des années. Dès lors qu'elle ne pourrait pas être d'un effet immédiat, elle prive mécaniquement le lanceur d'alerte de toute protection. » Comme nous l'avons dit lors des débats, l'arsenal juridique français est déjà très bien fourni en ce qui concerne la propriété intellectuelle, le secret médical, les secrets de fabrique ou encore la protection des secrets d'État, avec le fameux secret défense. Cette loi de transposition, voire de surtransposition, n'était donc pas indispensable

n'oseront plus divulguer d'informations et chacun s'imposera l'autocensure. Comme le souligne l'observatoire des médias Acrimed, ce texte s'inscrit dans une tendance durable, de la part des détenteurs du pouvoir économique, à mobiliser les ressources du droit pour dissuader les enquêtes portant sur la façon dont ils mènent leurs affaires et soustraire ainsi à l'attention du public des informations d'intérêt général. C'est une étape supplémentaire dans un travail de sophistication des outils juridiques permettant l'opacité, en lieu et place de la nécessaire transparence, et autorisant la définition de thèmes et d'objets considérés pouvant légalement faire l'objet d'investigations. Cette loi sera une arme au service des intérêts privés contre l'intérêt général.

Le secret et le mensonge sont incompatibles avec la démocratie. La différence entre démocratie et autocratie réside dans le rapport qu'elles entretiennent avec le secret. La démocratie est le gouvernement du pouvoir visible : le gouvernement public, en public. Dans l'autocratie le secret est la règle, tandis qu'en démocratie le secret est l'exception,

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, cette proposition de loi est un texte de défense de nos entreprises, donc de l'emploi de leurs salariés. Elle part d'un constat de bon sens : nous devons défendre les entreprises françaises contre l'espionnage industriel, je dirais même parfois le pillage de certaines de nos industries, qui s'est développé tout spécialement ces dernières années dans un contexte de mondialisation et de concurrence exacerbée entre les acteurs économiques. Il s'agit non pas d'un risque abstrait et futur, mais d'une réalité dont nous subissons les effets chaque jour. Ces pratiques contribuent à l'érosion de nos avantages compétitifs, à la perte de notre savoir-faire, au rachat de nos firmes et, finalement, à la perte d'emplois. Pendant ce temps, les pays qui sont les principaux partenaires économiques de l'Europe sont aussi souvent les premiers à prendre des mesures, afin de protéger leur savoir-faire commercial. La France était à la traîne. L'arsenal législatif européen et français n'est plus adapté à ces réalités. Il n'offrait pas même une définition unifiée du concept de secret des affaires, et cela a rendu notre économie vulnérable. Cette proposition de loi est donc bienvenue. Nos entreprises attendaient cette protection depuis plusieurs années. Le débat est ancien. Plusieurs tentatives ont eu lieu sous les gouvernements précédents, quelles que soient les majorités de gauche et de droite. Toutes ont échoué jusqu'au moment où la France a porté ce débat au niveau européen. La directive européenne que cette proposition de loi transpose a été en effet présentée sur l'initiative de la France par M. Cazeneuve, alors ministre délégué aux affaires européennes. La directive a été adoptée le 8 juin 2016 et votée par près de 80 % des parlementaires français au Parlement européen. Après de longs débats détaillés et approfondis, on doit se féliciter que le texte qui nous est présenté ait recueilli un très large accord sur l'essentiel. Protéger le savoir-faire de nos entreprises sans pour autant sacrifier la liberté de la presse : à première vue, ces objectifs peuvent paraître totalement contradictoires et opposés.

En réalité, les deux objectifs de défense des entreprises et de protection des journalistes et des lanceurs d'alerte m'apparaissent non pas concurrents, mais complémentaires. Il faut remercier les deux rapporteurs des commissions compétentes, particulièrement notre collègue Christophe-André Frassa, d'avoir su trouver un bon terrain d'entente. Le texte adopte une définition claire du secret des affaires, jusqu'alors fondé sur le droit commun de la responsabilité civile et la jurisprudence. Cela facilitera la tâche des entreprises et des juges. Il retient des critères cumulatifs particulièrement stricts, dans les termes de la directive. Il y avait débat sur la nature des informations protégées : fallait-il prendre en compte la valeur économique ou la valeur commerciale ? Toutes les données de nature économique détenues par une entreprise ne relèveront pas du secret des affaires. Seules le pourront celles qui font l'objet de mesures raisonnables de protection et qui revêtent une valeur commerciale effective ou potentielle pour son détenteur, lequel devra en apporter la preuve. Le texte apporte des garanties de procédure qui ont été renforcées durant les débats. Le dispositif a ainsi été étendu à l'ensemble des procédures devant les juridictions civiles, commerciales et administratives. Le Sénat avait souhaité créer une infraction spécifique sanctionnant l'atteinte au secret des affaires et l'espionnage économique. Nos collègues de l'Assemblée nationale penchaient plutôt le recours au droit commun- vol, recel, abus de confiance, intrusion dans un système informatique -ces qualifications leur paraissant suffisantes pour engager des poursuites. Sur ce point, je partage entièrement l'opinion de notre rapporteur : nous sommes dans une guerre économique ; un volet civil ne suffit pas, il faut un volet pénal. Faute de temps, nous n'avons pu procéder à toutes les consultations que nous aurions souhaité mener. la commission mixte paritaire, le président Philippe Bas a obtenu l'engagement de son homologue à l'Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, sur la poursuite de nos travaux sur cette question. Certains médias ont dénoncé ce texte comme instaurant une nouvelle forme de censure de la presse, pourtant abolie par la loi du 29 juillet 1881. Tel n'est pas le cas. Le texte comporte à ce sujet des garanties très claires et précises, sous le contrôle du juge. Le secret des affaires garanti par cette loi n'est pas absolu ; il est strictement encadré. Une entreprise ne pourra évidemment s'en prévaloir pour s'opposer aux enquêtes judiciaires ou administratives. Elle ne pourra pas davantage s'opposer à la révélation d'un secret des affaires, lorsque cette révélation est nécessaire pour l'exercice du droit syndical. Elle ne pourra pas obtenir de dommages et intérêts contre un salarié qui, de bonne foi et dans un but d'intérêt général, a porté à la connaissance d'un journaliste une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. En cas de révélation d'un secret des affaires, journalistes comme lanceurs d'alerte pourront toujours se prévaloir d'avoir agi dans le cadre de l'exercice légitime de leur liberté d'expression et d'information. Ces principes sont très clairement énoncés dans le texte qui vous est soumis. Le champ de la protection a d'ailleurs été élargi par la commission mixte paritaire par le rétablissement de la procédure d'amende civile, afin de répondre au risque de ce que l'on a appelé les « procédures bâillons Je persiste à penser, avec M. le rapporteur, que cette procédure n'était pas indispensable et qu'elle présente des risques d'inconstitutionnalité, que la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017 a mis à jour. À l'Assemblée nationale, vous avez annoncé, madame la garde des sceaux, que le Gouvernement avait décidé de confier à M. le député Gauvain et à M. le sénateur Frassa, rapporteur de la proposition de loi, une mission d'analyse des mesures de protection des entreprises françaises confrontées à des procédures judiciaires ou administratives de portée extraterritoriale. Vous avez évoqué, notamment, la loi de blocage de 1968. Je profite de ce débat pour vous demander si le Gouvernement entend prendre des initiatives à ce sujet au niveau européen. Alors que se met en place une guerre commerciale venant d'outre-Atlantique, l'Europe est-elle prête à réagir ? En conclusion, je voterai ce texte, avec les autres lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

le Défenseur des droits a recommandé l'abandon des dispositions de l'article 8 de ce projet de loi. Il se réfère notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire du 2 février du 2 février 2012, selon laquelle « l'effectivité du recours garantie par l'article 13 de la Convention européenne en cas de refoulement susceptible de faire naître un risque de traitements contraires à l'article 3, l'existence d'un recours de plein droit suspensif » pour motiver son avis. Or les modifications introduites par l'article 8 reviendraient à priver de caractère suspensif la plupart des recours introduits par des demandeurs d'asile en procédure accélérée, alors même que la réforme de 2015 avait consacré le caractère suspensif

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

8. En effet, le projet de loi prévoit que le droit au maintien sur le territoire, garantie introduite par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile prendra fin désormais à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et non plus à compter de la notification de la décision au demandeur.

ajouter que les dispositions prévues par cet alinéa vont à l'encontre de la notion de notification, qui impose un envoi, mais aussi une réception, qu'il faudrait par exemple attester par un recommandé. Cela constitue à notre avis un affaiblissement du droit de recours effectif

des sans-papiers qui, dans les faits, ne sont plus à la disposition des autorités françaises. Mes chers collègues, si vous voulez que le droit d'asile soit parfaitement défendu pour ceux qui l'obtiennent,

était susceptible de remettre en cause « l'effectivité de ce recours, laquelle suppose sa disponibilité et son accessibilité, non seulement en droit, mais aussi en pratique ». Une fois de plus, la volonté de réduire les délais va à l'encontre du droit à un recours effectif, principe auquel les auteurs de cet amendement sont attachés.

Cet amendement vise à supprimer un cas nouveau dans lequel le caractère suspensif du recours ne s'appliquerait pas : en cas de demande de réexamen jugée irrecevable. Outre que le recours suspensif doit demeurer le principe pour le demandeur d'asile, le CESEDA prévoit déjà que le recours suspensif ne s'applique pas en cas de demande de réexamen jugée irrecevable présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, ce qui devrait rassurer M. Karoutchi.

décision de rejet pour une demande examinée en procédure accélérée pour pays d'origine sûr, demande de réexamen ou menace à l'ordre public. En effet, ces exceptions reviendraient à couvrir un nombre considérable des décisions de l'OFII et donc à faire du caractère suspensif du recours un droit résiduel.

de supprimer la construction baroque que le Gouvernement a conçue pour essayer d'éviter les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme à la suite de la suppression

et de l'intégration est de coordonner et animer le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il prend ainsi en charge la gestion des entrées dans les centres d'hébergement et participe au dispositif du premier accueil des demandeurs d'asile. je l'ai fait remarquer hier encore, qu'il s'agisse de l'hébergement ou de l'interprétariat, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane restent préoccupantes, certainement plus qu'ailleurs. Si le raccourcissement des délais répond à une situation particulière, il est indispensable de veiller à ce que les droits des demandeurs d'asile soient préservés, et leur accueil dignement de l'article 8 , notre rapporteur a souhaité inclure des représentants des collectivités territoriales dans le conseil d'administration de l'OFII, afin de garantir une meilleure concertation avec les territoires. Eu égard aux situations spécifiques en matière d'asile et d'immigration que connaissent certains territoires ultramarins, en particulier la Guyane et Mayotte, les auteurs de cet amendement proposent que la composition de ce conseil d'administration assure une représentation des départements et collectivités d'outre-mer.

Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. L'article 9 du présent projet de loi porte excessivement atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs d'asile, dans la mesure où il contrevient à ce droit inconditionnel à l'accueil et au maintien en hébergement d'urgence de toutes les personnes au regard du seul critère de détresse. En effet, cet article vise à légaliser la circulaire du 12 décembre 2017, en prévoyant des modalités d'échange d'informations entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le service intégré d'accueil et d'orientation s'agissant des demandeurs d'asile et des personnes ayant obtenu une protection. Il s'agit de la mise en place d'un fichier recensant les personnes accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence, afin de connaître leur situation administrative- Dublin, fuite, débouté -, pour déterminer si elles ont toujours droit à cet hébergement. Ce dispositif inquiète, notamment, et à juste titre, les travailleurs sociaux, qui pourraient être sollicités en vue d'établir la liste des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale devant être transmise par le SIAO à l'OFII. Or, comme le Défenseur Or, comme le Défenseur des droits l'a souligné dans une de ses récentes décisions, les missions d'accompagnement des travailleurs sociaux sont difficilement compatibles avec des missions de sélection ou de contrôle. De fait, ces dispositions servent la politique du chiffre en matière d'expulsions et organisent la surveillance et le contrôle des migrants dès le début de leur parcours en France, au détriment de l'accueil et des droits fondamentaux des personnes.

il renforce le caractère directif du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, puisque le demandeur sera désormais orienté vers une région précise, où il sera tenu de résider. Le contrôle des autorités est intensifié, et de nouvelles hypothèses de retrait ou de suspension des conditions matérielles d'accueil sont prévues si l'étranger a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou s'il a quitté la région désignée par l'OFII sans en informer celui-ci. Le retrait de ces conditions matérielles d'accueil- hébergement ou allocation -est d'effet immédiat. Le Défenseur des droits estime que la mise en oeuvre du schéma national d'hébergement ne peut se réaliser que si elle est faite dans l'intérêt des demandeurs d'asile, sans que l'assignation à résidence aboutisse à un système de prérétention administrative, et qu'elle doit, en tout état de cause, s'accompagner d'une augmentation de l'offre des C'est ce qu'il préconisait déjà lors de la mise en place de ce schéma par la loi de 2015. Rappelons que, si la directive Accueil autorise les États à prendre de telles mesures, il ne s'agit que d'une possibilité. Son article 7 précise que « les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil Par ailleurs, si certaines améliorations ont été apportées au projet de loi, comme la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, le droit des demandeurs qui souhaitent être hébergés dans leur famille ou chez un tiers ne paraît pas expressément garanti. Or, en excluant du bénéfice des conditions matérielles d'accueil les demandeurs d'asile souhaitant être hébergés dans leur famille ou chez un tiers, le projet de loi va bien au-delà de ce qu'autorise la directive Accueil, qui n'a jamais exclu le principe de l'hébergement chez un particulier. Pour toutes ces raisons, nous nous inquiétons, comme d'ailleurs l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, de la porosité croissante entre l'accueil et la détention. Sous couvert d'un accueil encadré et efficace, cette politique migratoire organise la surveillance des personnes étrangères, des violations massives de leurs droits et, finalement, leur rejet.

leurs droits, d'un toit au-dessus de leur tête, pour ensuite entreprendre sereinement les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour. Pourtant, les mesures contenues dans l'article 9 ne sont pas satisfaisantes. rend plus coercitifs et directifs les dispositifs relatifs à l'hébergement prévus par le CESEDA : le demandeur d'asile sera orienté vers une région précise, où il sera obligé de résider. Par ailleurs, rien n'est prévu pour les requérants qui souhaitent être hébergés dans leur famille ou chez un tiers. Plus grave encore, cette fois sur le plan éthique : par cet article, entrerait dans le champ législatif l'inique circulaire Collomb du 12 décembre 2017. Rappelons que celle-ci prévoyait l'échange d'informations entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le service intégré d'accueil et d'orientation, afin de permettre la création d'un fichier recensant la situation administrative des exilés est de déceler ceux qui ne devraient plus bénéficier du droit à l'hébergement. De manière évidente, cet article contrevient au droit inconditionnel à l'accueil et au maintien en hébergement d'urgence des exilés en détresse

une de plus. Je veux parler de la formation linguistique du demandeur d'asile. Nous le savons, l'apprentissage du français est un vecteur essentiel d'autonomie pour le demandeur d'asile. La langue constitue une barrière ; elle rend les demandeurs d'asile dépendants des structures et des intervenants sociaux qui les accueillent.

Il s'agit d'une demande des associations qui oeuvrent au quotidien pour l'autonomie des demandeurs d'asile. La culture, l'éducation et le sport sont des vecteurs importants d'intégration et d'émancipation pour les nouveaux arrivants. Ils permettent de créer du lien social et d'apprendre la langue et la culture françaises dans un environnement diversifié et mixte.

L'article 9 du projet de loi réforme les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, comprenant les dispositifs d'hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile. Pour cela, il rend plus directif le schéma national d'accueil des demandeurs, qui qui déterminera désormais la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. Il soumet également l'octroi des conditions matérielles d'accueil à des conditions plus restrictives, telles que la résidence effective dans la région vers laquelle le demandeur a été orienté, ainsi que la bonne coopération avec les autorités françaises durant la procédure d'asile. Aujourd'hui, quelque 60 % des demandeurs d'asile sont concentrés dans

notamment le développement de campements insalubres se caractérisant par des conditions de vie précaires, qui ne manquent pas d'inquiéter les riverains. En conséquence, il serait souhaitable que la mise en oeuvre de l'hébergement directif se fasse vers des structures permettant un accompagnement effectif, décent et adapté à la vie privée et familiale de chacun. Il s'agit ici, tout simplement, de garantir aux demandeurs d'asile le respect de leur dignité. Toutefois, ces questions dépassent notre cadre national, car c'est l'Europe entière qui est touchée par la crise migratoire. Mardi dernier, à Berlin, le conseil des ministres franco-allemand, réunissant Emmanuel Macron et Angela Merkel, a mis en lumière la nécessité d'une réponse européenne commune à la question migratoire, afin que chacun

Pourtant, le Gouvernement entend renforcer ce caractère directif et coercitif, dans la mesure où le demandeur d'asile serait désormais orienté vers une région précise, où il serait obligé de résider.

Pour ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent la suppression de l'article 9, qui contrevient de manière évidente au droit inconditionnel à l'accueil et au maintien en hébergement d'urgence des exilés en détresse.

veut conserver l'orientation nationale des demandeurs d'asile, ce qui est une bonne chose, mais il supprime la garantie d'un hébergement. Cela revient à assumer l'idée que l'on enverra des demandeurs d'asile dans des régions qu'ils ne connaissent pas et où ils n'ont aucun contact, sans leur garantir un hébergement au bout. Il faut avoir à l'esprit, de surcroît, que le respect de cette orientation conditionne l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile. Il s'agit donc d'une question fondamentale. Imaginez un demandeur d'asile à qui l'on demanderait d'aller en Normandie,

Tout le dispositif proposé par le Gouvernement- l'orientation directive sans garantie d'hébergement, l'accord préalable de l'OFII pour sortir de la région, la multiplication des cas de retrait automatique des aides, etc. -revient à parquer les demandeurs d'asile et à faire peser sur eux la menace constante d'une suppression de toute aide matérielle. Non seulement l'hébergement doit rester la contrepartie de l'orientation directive, mais les schémas régionaux d'accueil doivent prendre en compte les situations personnelles et la vulnérabilité des personnes. Les conditions matérielles doivent pouvoir être sollicitées tout au long de la procédure et des prestations sociales et administratives minimales doivent être assurées dans

en tout cas avec une attention toute républicaine ! Alors ça ! Vous avez fait preuve, chers collègues, et vous ferez encore preuve dans les jours qui viennent d'une grande technicité.

J'ai tout entendu : l'orgueil d'être un pays attractif, la tradition d'accueil de la France, l'humanisme, les droits de l'homme, l'éthique, la nécessaire écoute, la prise en compte des persécutions, des souffrances- de toutes les souffrances. Je les ai toutes entendues ces souffrances, sauf une. Il existe une souffrance dont personne ne parle ici, c'est la souffrance du peuple français Le peuple français souffre de cette folle politique d'immigration, qui se traduit, chaque jour un peu plus, par une immigration non plus de peuplement, mais de remplacement,

57 % des Français refusent que de nouveaux bateaux puissent accoster dans notre pays. Vous refusez de l'entendre ! L'opinion publique,

a sa propre théorie. Nous l'avons entendu ici comme dans d'autres pays européens. Les propos sur le « grand remplacement » sont extrêmement choquants, parce qu'ils ne reflètent nullement la réalité de ce que vit notre pays, pays, parce que ce dont nous débattons aujourd'hui, mes chers collègues, c'est de l'avenir d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont dans l'obligation de quitter leur pays au risque de leur vie.

Monsieur le président, mes chers collègues, nous discutons de la politique de l'immigration et de l'asile, et il est parfaitement naturel que les points de vue s'opposent, parfois avec enthousiasme,

que, lorsque les choses ont été dites une fois, il peut être utile de les dire une seconde fois, mais les répéter dix ou quinze fois,

depuis plusieurs jours maintenant, nous n'arriverons pas au terme de cette discussion si nous n'assumons pas, en notre âme et conscience, la responsabilité de contenir ce débat, pour ce qui concerne le temps que nous lui consacrons, dans des limites raisonnables, et

Le scrutin est ouvert.

le demandeur d'asile peut demander à bénéficier des conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit. Aujourd'hui, il n'y a accès qu'en début de procédure. Or la situation des demandeurs d'asile peut évidemment évoluer